J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2021 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

sauvetage en mer (SNSM) des Sables-d'Olonne faisait naufrage, entraînant la disparition de trois sauveteurs. Ce drame avait ému la France entière, et le Président de la République s'était rendu sur place pour remettre la Légion d'honneur, à titre posthume, à ces « héros », pour citer ses propres termes.

La taxe sur l'aviation civile est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret ou de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) considère qu'une unité de trafic correspond à un passager ou à 100 kilogrammes de fret. Pourtant, le niveau de la taxe sur l'aviation civile ne respecte pas ce principe. En effet, un passager, soit une unité de trafic, paie entre 4,63 euros de taxe pour un vol intra-Union européenne et 8,32 euros pour toute autre destination, tandis qu'une tonne de fret, soit dix unités de trafic, est actuellement taxée à 1,37 euro. Cette absence de proportion équivaut à une niche fiscale hautement contestable, accordée au fret aérien sans justification. Dans un contexte de prise de conscience de l'empreinte carbone du transport aérien, et alors même que le transport de fret aérien alimente essentiellement la mainmise des GAFA sur le commerce en ligne, il serait à la fois logique et cohérent de remonter la taxe sur l'aviation civile.

d'atteindre la neutralité carbone du transport aérien. répondre à une exigence à la fois de justice et de protection environnementale en instaurant une progressivité de la taxe dite « Chirac », en fonction du type de billet.

comprenant l'augmentation des tarifs de l'écotaxe, l'ajout d'une tranche concernant l'aviation d'affaires et la modification du critère de destination, sur laquelle, je le rappelle, le Président de la République s'est lui-même engagé en juin dernier.

comme pour les passagers des véhicules domestiques. C'est sur cette base que nous avons calculé un forfait de 15 euros en classe économique et de 45 euros en classe supérieure pour un vol de moins de 2 200 kilomètres et respectivement de 30 euros et 90 euros pour un vol plus lointain.

Entre 2020 et 2021, le nombre de clients de ce secteur a connu une croissance de 50 %, et, selon un rapport de l'ONG Transport et environnement du 27 mai 2021, la pollution des jets privés a augmenté de près d'un tiers en quinze ans. Ce mode de transport est dix fois plus polluant qu'un avion de ligne et cinquante fois plus que le train.

alimentaires usagées. Même si ces matières premières permettent de produire des biocarburants avancés avec un impact environnemental réduit, les huiles alimentaires constituent un gisement très limité. Promouvoir leur utilisation pour l'aviation n'est donc pas souhaitable. En France, elles représentent un gisement de 50 000 tonnes par an, ce qui est très inférieur à la demande du secteur aérien. Par ailleurs, ce gisement est déjà mobilisé pour d'autres usages, notamment la production de biocarburant pour les transports terrestres.

l'exportation d'huiles usagées par les pays asiatiques entraînera un report de leur demande intérieure sur l'huile de palme, ce qui fera encore progresser la déforestation. Les auteurs de cet amendement proposent donc de ne pas définir d'objectif d'incorporation d'huiles alimentaires usagées et de graisses animales pour les carburéacteurs.

Cet amendement vise donc à rétablir, à partir de 2022, un tarif par hectolitre de nature à restaurer le caractère incitatif de la Tiruert et à soutenir l'incorporation de biodiesel dans les gazoles.

de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), à la discrétion du Gouvernement, activable par décret en fonction des coûts d'approvisionnement en gaz naturel. Cette baisse de taxe doit normalement permettre de faire face

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de taxe intérieure sur les produits énergétiques pour les paquebots de croisière. Il s'agit d'une niche fiscale nuisible pour le climat et génératrice d'externalités négatives fortes pour les riverains des ports, avec des incidences pour la santé publique et l'environnement.

Dans ce cadre, la suppression de la politique fiscale accommodante ou, pour le dire autrement, la suppression de la niche fiscale dont bénéficie le transport aérien, notamment le fret aérien, fortement émetteur de gaz à effet de serre, serait logique. Il y a, en l'occurrence, un véritable écart de concurrence entre les moyens de transport. Pourquoi donner à l'aviation cet avantage fiscal dont ne bénéficie pas, par exemple, le fret ferroviaire ? Je tiens à rappeler que les exonérations sur le kérosène représentent aujourd'hui 7 milliards d'euros. Gardons à l'esprit qu'il s'agit à l'évidence d'une injustice fiscale. Chaque fois que nous déposons cet amendement, on nous rétorque systématiquement que la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale de 1944 exempte de toute taxe les carburants d'aviation destinés aux vols internationaux. Toutefois, la directive 203/96 du Conseil prévoit que les États membres peuvent limiter son champ d'application aux transports internationaux et intracommunautaires, ce qui signifie donc que la taxation des seuls vols nationaux est bien possible et que rien ne s'oppose à ce que l'on rétablisse pour eux la TICPE.

Composantes essentielles de notre sécurité civile au sein des territoires, en particulier ruraux, les SDIS doivent être accompagnés dans leurs missions d'assistance et de secours aux personnes. Avec la multiplication des grands incendies pendant la période estivale, mais aussi d'autres défis tout le reste de l'année- catastrophes naturelles, sécurité et secours aux personnes -, les SDIS ont plus que jamais besoin de notre soutien. Aussi, afin de favoriser leur développement comme véritable socle de notre dispositif de secours, il est indispensable de faciliter leur organisation matérielle. Il est donc nécessaire qu'ils puissent orienter davantage leurs dépenses vers l'investissement et qu'ils bénéficient, à l'instar de nombreuses professions, de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). C'est pourquoi le présent amendement vise à exonérer les SDIS de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Quel est l'avis de la commission

ne prévoit pas d'exonération possible pour les services départementaux d'incendie et de secours. Malheureusement, c'est la même chose pour les forces armées, les forces de l'ordre ou les administrations.

Il s'agit d'un biocombustible liquide, ou biofioul, contenant jusqu'à 30 % d'esters méthyliques d'acides gras (F30). L'amendement vise à créer une nouvelle ligne à l'article 267 du code des douanes pour le F30 et à lui appliquer la même fiscalité que le fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible. Ainsi, la disposition proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l'année. Elle prend également en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés

L'objet du présent amendement est de reconnaître cette solution de rechange, qui est cohérente avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières au fioul 100 % fossile à partir du 1 juillet 2022. L'étude d'impact du décret d'interdiction souligne notamment que cette interdiction offre la possibilité d'installer des équipements alimentés en biocombustibles liquides, dès lors qu'ils respecteront le seuil. À cette fin, il convient de reconnaître la mise en place de ce processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un biocombustible en partie renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d'émissions de gaz à effet de serre.

en leur redonnant le surplus de recettes de TVA et de TICPE engrangé mécaniquement par l'État du fait des hausses des cours. La mise en oeuvre de cette TICPE flottante permettrait d'assurer de façon continue un lissage des effets de la hausse des prix sur le marché serait favorable à l'ensemble des consommateurs. Je pense qu'il est temps de prendre des mesures fortes pour défendre le pouvoir d'achat des ménages. La hausse des prix du pétrole ne doit pas conduire l'État à encaisser des recettes supplémentaires de TVA au détriment du pouvoir d'achat

nous pensons qu'il est davantage affecté par les politiques de dumping social exercées au sein de l'Union européenne que par la fiscalité écologique. Par ailleurs, d'autres pistes de soutien à nos PME de transport pourraient être envisagées Nous proposons donc de supprimer l'avantage fiscal aux entreprises étrangères qui viennent en France faire le plein, mais qui, dans le même temps, ne respectent pas les conditions d'emploi des salariés en matière de rémunération ou de coupure, par exemple.

dès 2022, une diminution du dégrèvement accordé au transport routier de marchandises de la TICPE sur le gazole et à placer ainsi, à terme, ce secteur polluant à un niveau de taxation équivalent à celui qui est acquitté par les automobilistes particuliers. Il est évident que la suppression des avantages fiscaux pour le diesel doit être accompagnée de mesures de compensation. Une telle disposition ne doit en aucun cas pénaliser les TPE et PME qui seront soumises aux nouveaux barèmes. Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

de brutalité. Les Français doivent savoir, notamment les trois millions de foyers qui se chauffent au gaz naturel, que les principaux pollueurs bénéficient d'une fiscalité huit fois inférieure.

des communes de Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses et Villejuif. Elle est aujourd'hui en grande difficulté en raison de l'augmentation des prix du gaz. Ce qui est le plus grand réseau de géothermie d'Europe

son équilibre économique. En effet, le gaz est utilisé par ce réseau de géothermie pour alimenter des chaufferies d'appoint nécessaires à la production de chaleur. Il y a deux tiers de géothermie et un tiers de gaz naturel pour ce réseau qui alimente l'équivalent de 36 000 logements. La hausse considérable des prix du gaz menace l'équilibre financier de la société, qui ne pourra y faire face et qui risque véritablement un dépôt de bilan. Cette situation a des conséquences pour les usagers. En outre, la hausse du prix sur ces usagers ne couvrira pas la hausse brutale du prix du gaz. Le lissage ne peut

concernant la part de gaz qui sert à produire de la chaleur, l'exonération n'est pas en vigueur. C'est pourquoi cet amendement tend à proposer une exonération sur la TICGN

naturel ce seul secteur poserait clairement la question de l'égalité de traitement vis-à-vis des autres secteurs qui subissent également l'augmentation des cours du gaz.

Cet amendement vise à soutenir le développement du biocarburant d'origine renouvelable en permettant une exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. Cette mesure s'inscrit en cohérence avec le projet de révision de la directive européenne sur la taxation de l'énergie (ETD), qui prévoit de distinguer clairement la fiscalité des carburants, selon qu'ils soient fossiles ou renouvelables.

Cet amendement vise à mettre en place une écocontribution, envisagée à 0,03 euro par unité, sur les produits en plastique ne pouvant démontrer l'existence d'une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à la situation actuelle et de cesser de taxer les gestionnaires des déchets, qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal-prix sur l'amont, au stade de la conception.

le plastique neuf, non indispensable et non recyclable. C'est un enjeu majeur, car près d'un tiers des déchets ménagers des Français sont composés de produits n'ayant pas de filière de recyclage, soit environ 200 kilogrammes par an et par habitant. Les mesures actuelles sont insuffisantes. Nous saluons le développement des filières à responsabilité élargie des producteurs. Cependant, 50 % des déchets faisant l'objet d'un stockage ne bénéficient toujours d'aucune de ces filières ou d'autres filières de recyclage. C'est d'autant plus problématique que cela rend impossible la division par deux du stockage prévu pour la croissance verte, afin de réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge. Aujourd'hui, la gestion de ces déchets est à la charge du contribuable. D'une part, les metteurs sur le marché des produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge ne contribuent pas à la gestion des déchets. Pis, ils ne sont pas incités à changer leurs pratiques et à se tourner vers l'économie circulaire. D'autre part, la collecte et le traitement de ces déchets issus du plastique, ainsi que le paiement de la TGAP sur ces opérations, sont à la charge des collectivités, ce qui se répercute

s'appliquerait à l'ensemble des « produits manufacturés » non couverts par une filière REP, à l'exception des produits alimentaires et énergétiques, cette notion demeurant toutefois très floue et juridiquement peu solide.

d'accompagnement à la réduction des déchets pour les entreprises produisant les produits manufacturés. Je note d'ailleurs que le Gouvernement a mobilisé 500 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour l'économie circulaire. Cette démarche, dans son esprit,

de jambons, ne sont pas recyclables. Les plastiques qui constituent les pots de yaourt sont en polystyrène : ils ne sont pas recyclables non plus. Certains pays

L'amendement n° I-717 tend à prévoir un mécanisme d'exception pour les petites entreprises. Les recettes financières ainsi créées pourraient être consacrées au développement de l'économie circulaire, mais aussi à l'accompagnement des politiques de réduction des déchets et d'écoconception des entreprises. À mon sens, rien ne vous empêche, chers collègues, de voter cet amendement.

La production et la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) constituent une solution de substitution au stockage, en valorisant énergétiquement des déchets qui ne peuvent être recyclés et en permettant ainsi la production d'une énergie locale. Cependant, la filière peine aujourd'hui à décoller et ne peut se développer sans aide. Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement soumises à la TGAP sur les déchets réceptionnés en entrée. Toutefois, la TGAP reste applicable aux refus issus d'unités de préparation de CSR, qui doivent être orientés en incinération ou en stockage. Une exonération de TGAP sur ces refus pourrait être un levier au développement de la filière. Quel

rectifié . On dénombre en France plus de 22 000 stations d'épuration urbaines de taille très diverses. La très grande majorité des stations- environ 18 000 -sont des petites stations d'une capacité inférieure à 2 000 équivalents-habitants, dotées souvent de technologies rustiques et peu énergivores. L'ensemble des stations d'épuration françaises produit environ 1 million de tonnes de boues, soit à peu près 7 à 8 millions de tonnes de matières brutes. La principale voie de valorisation et de traitement des boues urbaines est l'épandage agricole, qui concerne 44 % des boues. Depuis l'arrêté du 30 avril 2020, l'épandage des boues non hygiénisées a été interdit en France à cause du covid. Ainsi, de nombreuses collectivités chargées de l'assainissement ont été amenées à modifier en urgence le débouché de leurs boues d'épuration, pour s'orienter vers une filière hygiénisante ou vers l'élimination, avec, à la clé, de forts surcoûts, qui se reportent sur la facture des abonnés. Le présent amendement vise à exonérer de TGAP les collectivités qui ont dû modifier la filière de traitement, afin de faire face à la crise covid.

Pour autant, ils sont épargnés par des mécanismes financiers qui pourraient inciter à réduire leur utilisation. Les producteurs d'engrais sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes du fait des émissions suscitées par ce secteur, mais leur contribution reste infime, car les seuils d'émissions de polluants à partir desquelles les entreprises sont taxées sont beaucoup trop élevés. Par ailleurs, certains polluants majeurs sont exclus de cette taxe, comme l'ammoniac, qui constitue la matière première des engrais azotés. En 2016, les secteurs des produits chimiques, des engrais et des matières plastiques ont ainsi contribué seulement à hauteur de 6,7 millions d'euros, soit 0,09 % de leur valeur ajoutée. Le rapport de l'inspection générale des finances (IGF) de 2018 conclut au taux actuel de taxation, la TGAP n'est pas susceptible d'influencer les décisions d'investissement des industriels. Pourtant, les implications de la production d'engrais de synthèse sur la qualité de l'air et la crise climatique justifieraient une approche tournée

je veux mettre en avant une étude nationale menée par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air concernant l'impact sur cette dernière d'un certain nombre de

s'agit de compléter le dispositif prévu par le Gouvernement par un volet incitatif. Nous souhaitons créer une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif de réduction du stockage défendu par le Gouvernement, soit une division par deux des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010. mesure renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur en ce qui concerne l'élimination des déchets, en maintenant un signal-prix sur le stockage et l'incinération pour les collectivités qui n'ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts nécessaires.

Cet amendement vise à reporter l'augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Bien que la volonté de créer un signal-prix sur l'élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets.

Cet amendement tend à éviter que les collectivités ne soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le Gouvernement sur la publication des textes d'application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire, d'autant que cette sanction financière serait répercutée sur le contribuable local. Quel

lorsque les installations maximisent leurs performances environnementales ou que les collectivités sont parvenues à réduire leur flux de déchets mis en décharge ou à l'incinération.

pour les déchets non valorisables me paraît plus pertinente qu'une solution consistant à moduler les tarifs de TGAP en fonction des caractéristiques de l'installation de stockage et d'incinération de ces déchets, ou en fonction des performances des collectivités. En effet, les territoires et leurs collectivités n'ont pas forcément le choix des unités d'installation

Mme Viviane Malet. Les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution font face à des enjeux majeurs pour la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, sur le plan tant financier que technique. Le contexte de ces territoires conduit à ce que l'augmentation de la TGAP ne soit pas incitative, mais pénalise les budgets des collectivités, malgré les stratégies menées dans ce domaine. Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes réunionnais développent des projets visant à atteindre les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La réfaction demandée

Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraîne une baisse du rendement énergétique, faisant passer certaines installations sous le seuil de 65 %, qui permet de bénéficier d'une réfaction de TGAP. Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des événements ne relevant pas de leurs actions, il est proposé d'assouplir le calcul du rendement énergétique pour l'année 2021. Ainsi, les collectivités et les opérateurs concernés auraient la possibilité, soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d'état d'urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l'année précédente, ce qui permettrait d'éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l'année, y compris en situation normale.

La surveillance de la qualité de l'air est assurée par 19 associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA), disposant d'un réseau d'environ 650 stations de mesure réparties sur le territoire. Elles sont financées de manière tripartite par l'État, les collectivités territoriales et les entreprises, qui peuvent déduire des montants de taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux émissions polluantes polluantes (TGAP-Air) dont elles sont redevables les contributions qu'elles leur versent, dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Afin de compenser la baisse des contributions des entreprises consécutive à la crise sanitaire, la loi de finances pour 2021 a porté la subvention versée par l'État aux AASQA de 18 à 32 millions d'euros. une enveloppe de 23 millions d'euros, actant ainsi une augmentation de 5 millions d'euros du budget par rapport au niveau précédant la crise sanitaire. Toutefois, cette subvention de l'État ne résout pas à plus longue échéance la problématique du financement des AASQA, affectées par la diminution structurelle des contributions des entreprises. Pour faire face à cette érosion des ressources, le présent amendement vise à relever le plafond de déductibilité des contributions des entreprises de 171 000 euros à 250 000 euros et le taux maximum de déduction de 25 % à 50 %, afin d'inciter les entreprises à augmenter leurs versements. Une telle augmentation est indispensable pour permettre aux AASQA d'assumer leurs missions dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le contexte

La hausse du prix des carburants est la conséquence de trois facteurs : le coût du produit pétrolier, soumis à l'évolution du marché, le taux de marge des distributeurs ou des transporteurs et les taxes.

Ces hausses constituent une menace pour les ménages, notamment les plus précaires ; les classes populaires et moyennes ne peuvent pas continuer à payer le prix fort de la transition écologique. C'est pourquoi le présent amendement vise à exclure les impôts, les taxes, les droits et les prélèvements sur l'énergie de l'assiette de la TVA.

Selon les calculs de l'association UFC-Que Choisir, en 2018, les consommateurs ont payé en double taxation 1 milliard d'euros d'électricité, 200 millions d'euros de gaz et autant pour le fioul domestique. Sur une facture moyenne de chauffage,

exclure les taxes de la base d'imposition de la TVA serait contraire au droit européen, en particulier à l'article 78 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui a été transposé

du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable. La fourniture de chaleur, lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de solaire 50 % à partir de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d'énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid, en revanche, ne sont pas soumis au même régime. Pourtant, la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid. Les étés seront de plus en plus caniculaires et, en conséquence, l'utilisation des climatiseurs va augmenter. La production de froid renouvelable, composante importante et méconnue des énergies renouvelables, est indispensable pour remplacer à terme l'ensemble des climatiseurs dans le tertiaire et l'habitat individuel ou collectif, qui sont d'importants consommateurs d'électricité et qui accentuent la création d'îlots de chaleur urbains. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le sud de la France, où les besoins de refroidissement augmentent chaque année. Dotée d'une très grande efficacité énergétique, la production de froid renouvelable est l'un des atouts majeurs de la géothermie, sous toutes ses formes,

à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsion de concurrence. La précision relative au chauffage urbain exclut d'office la fourniture des réseaux de froid, qu'ils soient

L'objectif de la France est de parvenir à en équiper 9,3 millions de foyers d'ici à 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a également instauré un objectif de baisse de 50 % des émissions de particules fines entre 2020 et 2030 dans les territoires couverts par un plan de protection de l'atmosphère, Le plan d'action pour un chauffage au bois domestique performant, publié par le Gouvernement en juillet 2021, permettra, d'ici à 2030, de réduire de 50 % les émissions de polluants du chauffage au bois domestique. Il fixe comme objectifs l'acquisition d'appareils performants, la structuration du marché

de qualité permettra de diviser par dix les émissions de particules fines des appareils de chauffage d'ici à 2030. Outre la diminution d'émissions de polluants, un bois sec permet un meilleur rendement qu'un bois humide. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée. Le présent amendement vise donc à appliquer le taux de TVA réduit à 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé et présentant un taux d'humidité inférieur à 23 %.

Il s'agit d'appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié attestant son caractère durable et local. Cette mesure concerne de nombreux secteurs : Bois

tous les sylviculteurs et exploitants forestiers à utiliser des procédés permettant de tirer le meilleur parti de la production forestière.

particulier, de la façon de brûler le bois ? La cheminée ouverte, le poêle, l'insert ont des degrés extraordinairement variés de performance énergétique.

Cet amendement vise à contrer l'effet des hausses de prix des énergies et des carburants constatées ces derniers mois : pour le gaz, l'augmentation est de 70 % depuis le début de l'année

Pour un ménage moyen utilisant ces énergies et carburants, selon le mix utilisé, le surplus sur la facture annuelle peut aller de 230 euros, soit une augmentation de 8,3 %, à 807 euros, soit une hausse de 27 %. Afin de limiter ces hausses de prix qui risquent de se révéler insupportables pour une partie de nos concitoyens, l'amendement tend à supprimer la « taxe sur la taxe

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement fait partie d'une série d'amendements du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain qui ont pour objet d'inscrire dans la loi des mesures soutenant le pouvoir d'achat des Français face à l'augmentation des prix de l'énergie. Aujourd'hui, la hausse des prix des carburants a de fortes incidences sur le pouvoir d'achat des Français, notamment de ceux qui résident loin des villes et des transports en commun. Le dispositif est certes coûteux pour les finances publiques. Mais, en 2018, au moment de la crise des gilets jaunes, le Gouvernement n'a pas pris de mesures ambitieuses dès le début de la crise, ce qui nous a coûté très cher. Aider les Français maintenant en leur rendant un peu de pouvoir d'achat reviendrait moins cher à la collectivité. Les mesures permanentes sont incompréhensibles, aujourd'hui où s'exprime une forte demande de justice sociale. Aussi, cet amendement vise à baisser la TVA sur la consommation de carburants à 5,5 %, jusqu'au 1 juillet 2022.

tous les ménages au regard de la préoccupation qui est la vôtre et la nôtre, sans prendre aucunement en compte les conditions de ressources. Enfin, d'une certaine manière,

Le gaz vert doit jouer son rôle pour atteindre les objectifs climatiques de la France. Le présent amendement a pour objet, sans surcoût pour les finances publiques ni pour le consommateur, un mécanisme territorial efficace visant à développer la production de gaz vert, en l'associant à la construction de nouveaux bâtiments. Afin de contribuer à la bascule du parc immobilier vers l'excellence environnementale et les énergies renouvelables avec un coût maîtrisé de la construction, cet amendement tend en effet à créer un mécanisme vertueux et facultatif de financement de la production de gaz vert qui ne pèse pas sur les finances publiques nationales ou locales qui ne renchérit pas, pour le promoteur comme pour l'acquéreur du bâtiment, les coûts de construction, qui sont la cible de la nouvelle réglementation environnementale, dite « RE2020 ». À l'occasion de la construction d'un bâtiment neuf soumis à la RE2020, le maître d'ouvrage aura la possibilité de choisir d'alimenter le bâtiment en gaz, en acquittant un prélèvement libératoire au conseil régional. Le montant correspondant sera ensuite versé au profit de la production du gaz vert nécessaire pour alimenter le bâtiment pendant les quinze premières années, en réponse aux exigences réglementaires, soit la durée de vie d'un équipement de production d'énergie renouvelable. L'amendement vise donc cette nouvelle compétence du conseil régional pour financer volontairement de nouvelles installations de production de gaz vert, par un prélèvement libératoire des maîtres d'ouvrage souhaitant offrir à leurs clients un chauffage au gaz vert vertueux et local.

aux promoteurs, puisque le prélèvement libératoire serait une action volontariste versée aux régions pour développer ce gaz vert. Enfin, notre proposition est sérieuse,

tendent à créer un prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz, dont le produit a pour objet de soutenir la production de biogaz. Celui-ci serait dû par les maîtres d'ouvrage des bâtiments neufs

Je dois aussi préciser que le verdissement du gaz est déjà encouragé par la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel qui a été introduite depuis le début de l'année, notamment lorsque le biogaz est injecté

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels qui sont des composés organiques ou métalliques susceptibles d'avoir une action toxique pour l'homme, mais aussi pour les organismes aquatiques, y compris à des concentrations très faibles dans l'eau. L'Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus de 20 000 en mai 2018 dans le règlement Reach, et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels. Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments et produits d'hygiène corporelle et domestique ou encore dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe, qui nécessite des actions préventives et curatives. Je pense à un encouragement à l'écoconception pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes ; à des des actions de réduction de l'utilisation des produits contenant ces micropolluants par de la communication auprès des consommateurs, mais aussi avec un signal-prix ; enfin, à des actions de prévention des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l'eau.

Les dispositifs de soutien financier existants, notamment les agences de l'eau et quelques responsabilités élargies du producteur (REP), qui ne sont concernées qu'à la marge, ne couvrent pas ces actions à grande échelle. s'agit aujourd'hui encore souvent d'actions menées à titre expérimental et qu'il va maintenant falloir généraliser au niveau national. Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d'ores et déjà existantes au niveau français et européen.

qui s'apparente à une taxe à la consommation, puisqu'elle représenterait entre 0,5 % et 1,5 % du prix des produits.

ce qui paraît plus logique. Il faudrait prendre le pari d'associer les industriels et les fabricants, plutôt que de laisser à la seule charge du consommateur

nitrates et les pesticides. L'objet de cet amendement est d'inclure l'azote de synthèse dans l'assiette de la redevance pollution diffuse dont doivent s'acquitter les agriculteurs. Selon la direction générale du Trésor, « en accroissant le prix relatif des engrais, la taxe serait susceptible d'orienter les comportements vers des pratiques économes en intrants et donc moins moins polluantes ». La mise en place d'une redevance sur le recours aux engrais azotés de synthèse en complément d'une politique de soutien au développement de l'agriculture biologique a montré des résultats significatifs sur la réduction des engrais chimiques en Autriche. Pour soutenir la transition agroécologique et répondre aux enjeux de justice sociale, les recettes d'une telle redevance doivent être entièrement réaffectées aux agricultrices et agriculteurs.

la production de légumes de contre-saison bénéficie d'une aide d'environ 25 000 euros par hectare tous les ans, alors que celle-ci était auparavant plafonnée à 20 000 euros tous les trois ans. Ce déplafonnement, qui profite aux plus grandes structures, entre en contradiction avec l'engagement du Gouvernement d'accompagner les filières pour les aider à sortir de leur dépendance aux niches fiscales défavorables à l'environnement. L'argent public, rare dans cette filière, doit être redirigé vers la sortie du chauffage et l'investissement dans des techniques de substitution au chauffage pour produire des légumes sur nos territoires- pense aux serres froides ou à l'isolation des serres -, en adéquation avec les aspirations des citoyennes et des citoyens. Pour les professions agricoles, dont les serristes, il existe un remboursement partiel de TICGN. Le montant du remboursement correspond à la différence entre le taux nominal de TICGN et un montant de taxe restant à la charge des agriculteurs, fixé à 0,54 euro par mégawattheure, taux minimum prévu par la directive